L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, dont le Sénat est saisi en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à la motion n° 4738 tendant au renvoi en commission de l'article 1.

Monge, pour la motion. L'article 1 du projet de loi vise à supprimer plusieurs régimes spéciaux ou autonomes. En réalité, les régimes spéciaux concernent non pas l'ensemble des salariés de ces branches, mais uniquement ceux qui ont les conditions de travail les plus dures.

en 2019, d'environ 6 %. Mettre fin aux régimes spéciaux et autonomes sous prétexte d'équité et de supposée universalité est une diversion visant à faire oublier que tout le monde pâtira du report de l'âge légal de départ à la retraite. Les régimes d'EDF et de la RATP, par exemple, prévoient de meilleures anticipations de départ et une meilleure prise en compte de la pénibilité.

de catégorie active, donc d'exposition à ces risques et facteurs de pénibilité, ils peuvent partir à 57 ans et, demain, à 59 ans. Nous n'avons pas eu le temps de débusquer en quoi ils seraient des privilégiés. La justice sociale et l'équité voudraient que l'on applique ces mesures sérieuses de prise en compte de la pénibilité à tous les travailleurs accomplissant des travaux pénibles, plutôt que de niveler par le bas,

Le groupe écologiste estime donc que le sujet des régimes spéciaux et de son impact sur la vie de milliers de travailleurs mérite, au préalable, un débat en commission

pour diviser les Français et faire passer la retraite par points. Monsieur le ministre, c'est un comble aujourd'hui de vous entendre vanter le régime par répartition, alors que vous vouliez l'abattre voilà à peine quatre ans. Vous entendez mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte de renforcer la justice sociale entre les futurs retraités. Vous allez plus loin et vous proposez des mesures plus dures que ne l'avait fait Nicolas Sarkozy Sarkozy en son temps. Les régimes spéciaux accordent des compensations à des travailleurs exerçant des métiers pénibles, qui exigent des astreintes fréquentes et entraînent une usure physique. Nous nous opposons à leur suppression injuste. Il faudrait que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles ces métiers ne nécessitent pas de mesures spécifiques d'aménagement des carrières, comme la possibilité d'anticiper les départs à la retraite afin de mieux prendre en compte la pénibilité. la pénibilité. Dans ces secteurs en effet, les travailleurs ont une espérance de vie souvent inférieure à celle de la moyenne des salariés. Nous souhaitons le maintien du modèle social actuel. Les régimes spéciaux ne sont pas des privilèges. Ambroise Croizat parlait d'ailleurs de « conquis sociaux ». Au lieu de fermer le régime de la RATP, des électriciens et des gaziers, de la Banque de France, du Conseil économique, il faudrait généraliser ces compensations à l'ensemble des travailleurs qui accomplissent des travaux pénibles. Notre groupe souhaite supprimer l'article 1, qui ferme des régimes spéciaux

une fois de plus, nous vous demandons l'avis du Conseil d'État que vous nous cachez soigneusement explication de vote. Monsieur le ministre, les régimes spéciaux constituent selon vous des privilèges, alors qu'ils ont été pionniers en matière de droits à la retraite. Ils ont été mis en place en raison de l'organisation et de la nature du travail dans les différents secteurs et sont le fruit d'une véritable conquête sociale, qui s'est construite au fil des décennies. Ces régimes fonctionnent, en outre, sur la base d'une solidarité restreinte à une profession.

gains escomptés par la suppression de ces régimes seront au regard des problèmes dont on parle. Il ne s'agit pas davantage d'une question de justice sociale : on ne fait jamais de justice sociale en tirant quelques dizaines de milliers de travailleurs supplémentaires vers le bas. le ministre, c'est qu'en vous attaquant à ces régimes spéciaux vous voulez continuer à démanteler des services publics dont nous avons absolument besoin pour relever le pays et le sortir de la crise actuelle. D'ailleurs, dans les secteurs concernés,

pose n'est pas une question de justice. Vous allez porter un coup aux capacités de reconstruction de nos services publics, dont nous avons besoin pour la transition écologique et la réindustrialisation du pays. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann,

mais surtout ni de gauche, qui menace de le faire. Quel est l'intérêt de supprimer des régimes autonomes tels que celui des gaziers ou des clercs de notaire, qui ne demandent rien à personne ? l'intérêt de vouloir rompre un contrat avec des agents de catégorie active de la RATP qui, de toute façon, ne prennent pas leur retraite à 52 ans, mais au minimum quatre ou cinq ans plus tard ? Quel est l'intérêt de verser au régime général des milliers de salariés,

en mettant fin aux privilèges inconsidérés d'une toute petite minorité qui se gaverait, au détriment de la grande majorité des salariés. Quelle est la réalité

600 000 personnes en invalidité bénéficient d'un régime général qui n'est pas le régime de base. Finalement, ce sont près de 40 % des assurés sociaux qui bénéficient d'un régime différent, hors fonctionnaires d'État. La réalité de la situation des retraites

moins de 1 % de la population active et vous en faites des boucs émissaires qui seraient à l'origine de tous les maux. Ce dont il devrait être question aujourd'hui, c'est précisément d'élargir ce que nous considérons en effet comme des régimes pionniers. régime de ce salarié de la RATP, dont il est question ces jours-ci et qui a été exposé à de l'amiante dans son travail d'électricien, aux

participe à l'attractivité des professions à l'heure d'une crise inédite en la matière. Le Gouvernement mobilise le principe de justice afin de justifier leur fermeture, mais votre chemin pour la justice est le nivellement par le bas et la diffusion dans tous les secteurs de la crise du travail et de l'attractivité.

pour diviser et faire diversion aux reculs que vous voulez appliquer ! Quant aux régimes autonomes, ce sont des régimes qui surcotisent pour des prestations plus généreuses que les autres régimes et sans subvention publique d'équilibre. Alors, que leur reproche-t-on ? De s'exclure de la solidarité inter-régimes ?

Je lisais récemment dans une excellente revue,, que les régimes spéciaux représentaient moins de 3,5 % de l'ensemble des cotisants de France et qu'ils ne pesaient pas tous le même poids. Les danseurs de l'Opéra de Paris ne sont que 168 et, si j'ai bien compris, vous n'allez pas leur imposer de danser jusqu'à 64 ans

mettent en péril l'ensemble du système. Bruno Le Maire a d'ailleurs déclaré : « C'est moins un problème financier qu'un problème d'équité. » L'équité, c'est une vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste. Mes chers collègues, il n'est pas juste de niveler par le bas je voudrais savoir ce que dit la note de synthèse du Conseil d'État sur ce sujet, car il ne s'agit pas d'un problème financier.

Aujourd'hui, vous nous proposez de supprimer des régimes spéciaux qui tiennent compte de cette pénibilité. Vous nous proposez l'alignement par le bas des régimes spéciaux qui prennent en compte, branche par branche, la pénibilité d'un certain nombre de métiers. Dans ces régimes spéciaux, les cotisations des salariés sont souvent supérieures à celles du régime général. Je pense en particulier au régime des industries électriques et gazières

Il faut dire la vérité aux Français : cette remise en cause des régimes spéciaux ne concerne pas l'ensemble des salariés du secteur qui seraient des privilégiés, comme cela a été avancé, mais uniquement celles et ceux qui ont les conditions de travail les plus difficiles. Je le redis, la création de ces régimes

Face à cela, il est nécessaire, une nouvelle fois, de rappeler quelques faits. Premièrement, les régimes spéciaux représentent moins de 3,5 % de l'ensemble des cotisants en France. Heureusement, votre stratégie d'accabler une minorité pour recevoir l'assentiment de l'opinion publique ne semble pas fonctionner. Deuxièmement, les régimes spéciaux ne sont pas une exception française, loin de là.

Alors que nous devrions défendre collectivement un projet d'amélioration de notre modèle social qui prenne en compte le quotidien des individus et la pénibilité de chaque profession, vous faites le choix de vous attaquer à des régimes qui étaient précurseurs par une juste appréhension du travail et de ses effets sur les travailleurs. Comme cela a été dit, il ne faut pas oublier que, lors de la création du régime général en 1945, les régimes existants, notamment celui des cheminots, ont été maintenus, car ils apparaissaient comme un horizon à atteindre pour le régime général. Nous reviendrons longuement sur la question de la pénibilité lors de nos débats, mais je pense que l'adoption de l'article 1 représenterait déjà une première atteinte particulièrement regrettable à notre système de protection sociale et illustrerait le manque de considération envers ces professions pénibles au quotidien. Pour éviter de nombreux pas en arrière et une atteinte aux fondements

Chacun voit bien qu'il est mis à mal, puisque les organisations syndicales s'opposent unanimement à ce texte. Deuxièmement, le principe du respect des engagements pris.

Aux Antilles, territoire à vocation agricole, les agriculteurs et leurs proches sont victimes des pesticides, en particulier du chlordécone. Ils souffrent de cancers. Vous avez pourtant réintroduit les néonicotinoïdes, il faut le savoir ! Dans le même temps, par incohérence ou provocation, vous avez supprimé

Cette suppression relève d'une logique, celle du Président de la République qui « n'adore pas ce mot de pénibilité, parce qu'il donne le sentiment que le travail serait pénible ». C'est ce qui a amené son gouvernement à vider de sa substance le compte professionnel de prévention, créé en 2015, en supprimant dès 2017 les quatre critères principaux qui permettaient aux salariés qui effectuent des travaux pénibles de cumuler des points pour partir à la retraite de manière anticipée. C'est la même logique qui prévaut avec cet article sur les régimes spéciaux. Vous choisissez un nivellement par le bas, alors que la justice et l'équité voudraient non seulement qu'on les conserve, mais surtout que l'on s'en inspire pour prendre en compte les difficultés de nombreux métiers. Oui, monsieur le ministre, mes chers collègues, porter des charges lourdes, travailler en horaires décalés, subir des vibrations mécaniques, travailler dans un environnement chimique dangereux, soulever des malades, tout cela est pénible. Ces régimes sont le fruit de conquêtes sociales par les travailleurs concernés et leurs organisations syndicales. C'est le fruit d'un compromis social. Notre conception de la relation au travail diffère de la vôtre. Nous considérons que la pénibilité existe, qu'elle pèse sur la santé des salariés et qu'elle doit se traduire par des gains en espérance de vie à la retraite en bonne santé, donc par un départ anticipé. C'est là de votre part une mesure de diversion, s'appuyant sur un postulat faux : l'opinion publique serait favorable à la suppression de ces régimes spéciaux. C'est une mesure de diversion et de division des salariés, car vous laissez croire que ceux qui bénéficient de ces conditions seraient des privilégiés, alors qu'en fait, comme tous les autres, ils subiront votre réforme

Vous voulez tout simplement appliquer aux régimes spéciaux les mêmes dispositions et les intégrer au régime général dans le cadre d'une réforme profondément injuste et brutale. Comme vous faites une réforme des retraites injuste qui frappera durement l'ensemble des Français, vous avez voulu détourner leur attention, en cherchant des boucs émissaires. Fidèles à vos penchants sarkozystes, c'est sur ce qu'on appelle les régimes spéciaux que vous avez choisi de vous acharner. Vous allez nous chanter la ritournelle habituelle et faire passer des règles dérogatoires pour des privilèges. Vous allez essayer de diviser les salariés de ce pays et plus généralement l'ensemble des Français. Vous allez nous parler du chauffeur de bus de la RATP et nous demander

qui ont été créés pour mieux compenser la pénibilité de certains métiers. Les régimes spéciaux sont non pas des privilèges, mais la juste compensation des contraintes du travail- travail de nuit, de week-end ou en sous-sol, horaires décalés, exposition à des risques chimiques,

la manutention manuelle des charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux risques chimiques. Une entrée en matière de mépris pour ceux qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. De plus, vous choisissez de supprimer certains régimes : la RATP,

Diviser pour éviter de parler des vraies inégalités, des vrais privilèges, des profits records, des profiteurs de crise. Diviser pour éviter de parler de justice sociale et d'équité, parce que vous n'aimez pas

Jean-Luc Fichet, sur l'article. Le Président Macron a supprimé des critères de pénibilité, en expliquant qu'il ne fallait pas donner le sentiment que le travail était pénible. En visitant le marché de Rungis, le président a peut-être- je dis bien, peut-être -entendu que les horaires, les charges lourdes, le stress, les troubles musculo-squelettiques, la charge mentale sont autant de raisons qui rendent les métiers pénibles, difficiles et peu attractifs.

sur l'article. Monsieur le ministre, par cet article, vous comptez mettre fin à la plupart des régimes spéciaux que notre système de retraite permet actuellement. Ces régimes constituent, selon vous, une dépense exagérée qui ne serait plus soutenable par notre système de retraite. En réalité, et vous le savez, les dépenses liées aux régimes spéciaux demeurent contenues en proportion des recettes totales de cotisations sociales. Plus encore, ces régimes permettent à des secteurs et à des cadres d'emploi de rester attractifs là où la main-d'oeuvre, pourtant essentielle, peine à être trouvée. Par ailleurs, vous préservez la faculté pour les hauts fonctionnaires de cotiser, donc de bonifier leur future retraite sans exercer la mission de service public en rapport avec cette retraite future- ce n'est pas un regret de ma part, bien au contraire.

Plus encore, monsieur le ministre, au-delà de ceux qui sont directement concernés par les régimes spéciaux, les Français ne veulent pas de votre réforme. Écoutez-les

C'est tout simplement la prise en compte de la dureté du travail, ce que l'on appelle maintenant pénibilité. Oui, certains métiers sont durs, abîment. Finalement, avons-nous abandonné l'idée même de progrès social ? Oui, j'ai bien dit progrès, ce n'est pas un gros mot : le progrès, c'est un avenir qui donne envie.

regard de toute la richesse produite dans notre pays, d'autres financements sont largement possibles. Voilà le vrai défi que ce texte devrait relever

est étonnante : on aurait pu débattre du rétablissement d'un certain nombre de facteurs de pénibilité au travail, on aurait pu débattre de progrès social ... Non ! En réalité, la ficelle est un peu grosse. Personne n'est dupe de cette tentative de diversion. Vous voulez monter les Français les uns contre les autres, mais vous n'y arriverez pas. Il n'y a aucune justice sociale, aucun progrès social dans le recul des droits des travailleurs. Personne ne souhaite niveler par le bas les conditions de travail. Vous ne parviendrez pas à briser l'union de tous les travailleurs contre votre projet de réforme. Cela a été dit, la particularité des régimes spéciaux ne vient pas de nulle part. Elle est le fruit d'une histoire, l'histoire sociale de notre pays, de notre République- parce que, oui, la République française est sociale. Justement, où sont les défenseurs de ce roman national, des valeurs de notre République ? Où sont celles et ceux qui n'ont de cesse de défendre l'universalisme, ce phare que devraient être la France et son modèle, celles et ceux qui ont la République à la bouche, mais uniquement pour nous diviser ? Nous sommes face à une crise du travail, de l'emploi de l'attractivité d'un certain nombre de métiers, qui met notamment à mal nos services publics. Votre engouement à détériorer en permanence les conditions et statuts de celles et ceux qui portent notre société, les essentiels, les premiers de cordée met à mal notre société et notre République. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, comme agriculteur, je suis rompu à des conditions de travail difficiles. Je crois pouvoir en parler.

qui l'avez faite ainsi ! J'ai envie de vous parler de ce régime spécial de la RATP, avec ses horaires atypiques, la fréquence des astreintes, l'usure physique,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le système de retraite est un ensemble complexe, qui produit de multiples interactions. Dès lors que l'on modifie l'un des éléments, celui-ci interagit avec d'autres, générant des effets induits, qu'il est important de discerner.

Nous abordons l'article qui supprime certains régimes spéciaux sous un angle budgétaire, sans nous soucier d'une vision globale sur ces régimes et des conséquences qui découleront de leur suppression.

national. Ils sont souvent discrédités et jetés en pâture à l'opinion, sans tenir compte de l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exercent les professions concernées, de leurs contraintes particulières, certes, mais aussi de l'ambition en 1945, il fallait reconstruire, relever les défis et mobiliser l'ensemble des acteurs et des citoyens. En 2023, nous avons l'immense défi de la transition énergétique, du développement des transports collectifs, énergies et mobilités. Tels sont les enjeux pour lesquels il faut désormais une ambition politique. Cette ambition ne pourra jamais être atteinte en stigmatisant ceux qui doivent en être les acteurs.

monsieur le rapporteur, très factuel : la majorité sénatoriale est constante dans ses positions. Voilà quatre ans que nous présentons un projet de réforme qui prend en compte une convergence des régimes spéciaux.

que l'ensemble des salariés voient les conditions d'exercice de leurs activités prises en compte de la même manière. La pénibilité, l'exposition à l'usure doivent être mesurées de la même façon, dans une logique d'effectivité des conditions d'exercice plutôt que dans une logique de statut. En effet, derrière une logique de statut, il peut y avoir des inégalités et, derrière un même statut,

d'avancer sur la prise en compte des critères ergonomiques comme sur l'amélioration du compte professionnel de prévention et, ainsi, de faire en sorte que les salariés et, au-delà, l'ensemble des travailleurs exposés à des conditions d'exercice difficiles soient mieux protégés. Nous avons fait le choix de proposer au Parlement la fermeture du régime d'assurance vieillesse uniquement pour cinq régimes spéciaux et de conserver tout particulièrement les avantages et conditions

dès lors que l'on retire les subventions spécifiques versées par l'État à certains régimes- par exemple, la RATP -ou des contributions ayant un caractère fiscal payées sur la facture de chacun des consommateurs- je pense aux IEG. Nous avons un devoir de responsabilité par rapport au coût pour la collectivité que représentent aujourd'hui des régimes qui, par leur logique de statut, entretiennent des iniquités, alors même qu'ils sont coûteux pour l'ensemble des contribuables. Tout cela n'est évidemment pas légitime. La seule question, derrière le financement des régimes spéciaux,

interventions : s'il existe une difficulté ou une forme d'iniquité- c'est peut-être, d'ailleurs, une façon de la reconnaître -, il faudrait que l'ensemble de celles et de ceux qui exercent des métiers identiques ou proches puissent bénéficier des mêmes conditions. J'ai notamment entendu que les agents de conduite des métros et des bus d'autres communes que celles qui sont couvertes par la RATP devraient pouvoir bénéficier des mêmes conditions de départ anticipé. Souvent, cette solution nous est proposée au nom du pragmatisme. C'est la démonstration que le pragmatisme et le réalisme ne font pas toujours bon ménage, en tout état de cause qu'ils ne sont pas synonymes ! En effet, une telle mesure aurait un coût absolument

n'ont pas de caractère public : seuls un certain nombre de parlementaires, du fait de leurs prérogatives de contrôle et d'évaluation, peuvent y avoir accès, s'ils le souhaitent et dans des conditions déterminées par la loi, mais aussi par le secrétariat général du Gouvernement. Je

Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 36 de notre règlement. Monsieur le ministre, vous le savez, nos travaux sont extrêmement suivis. D'ailleurs, les salariés des industries électriques et gazières ont décidé,

dès hier, procédé à des centaines de distributions d'électricité à celles et ceux qui en avaient été privés ou ont basculé les artisans, commerçants ou petites collectivités au tarif zéro. Ils se rappellent, d'ailleurs,

soit élargie à l'ensemble des intervenants. Je le dis très amicalement, l'intervention de Mme la rapporteure générale, qui s'adresse à une partie de l'hémicycle en lui posant des questions,

sollicitons une suspension de séance de quelques minutes pour réorganiser les dossiers de séance à la suite de nombreuses erreurs matérielles dans l'ordre des signataires des amendements. Acte vous est

L'indexation sur les prix fait donc basculer une grande partie des retraités dans la pauvreté et dans la dépendance aux aides sociales. C'est pourquoi il est absolument urgent d'amorcer dès maintenant un retour pour toutes et tous à l'indexation sur les salaires. Cela constitue une condition de la pérennité du système par répartition.

ambitieuses et sérieuses de prise en compte de la pénibilité à tous les travailleurs de toutes les branches qui accomplissent des travaux pénibles ou qui sont exposés à des facteurs de pénibilité, plutôt que de niveler les droits sociaux par le bas. La vraie question

La suppression de ces régimes spéciaux constitue une stratégie supplémentaire du Gouvernement pour faire oublier le principal : le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ce gouvernement est prêt à toutes les manoeuvres pour opposer les Français les uns aux autres. Les régimes spéciaux sont stigmatisés pour pouvoir niveler par le bas les droits à la retraite. Le but de ce gouvernement est clair : fissurer le front uni qui se dresse contre cette réforme injuste. Cette stigmatisation est d'autant plus injuste que les régimes spéciaux concernent non pas l'ensemble des salariés de ces professions, mais seuls ceux qui occupent des fonctions impliquant des conditions de travail difficiles. À titre d'exemple, seuls 5 % des salariés de la RATP sont concernés par son régime spécial.

n'y a là rien d'étonnant : cette réforme injuste s'inscrit dans la continuité de la politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017. La pénibilité et la souffrance au travail qui touchent les salariés sont complètement ignorées par ce gouvernement. République avait ainsi supprimé quatre critères de pénibilité en 2017 : les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les manipulations de charges lourdes et les agents chimiques dangereux. Et voilà que le Gouvernement veut maintenant supprimer ce qu'il reste de droits aux salariés qui travaillent dans des conditions difficiles

ceux qui bénéficient des superprofits et de la rente sont exemptés. Pourtant, ce sont bel et bien celles et ceux qui travaillent qui savent ce qu'est la valeur du travail une valeur non pas morale, mais économique et marchande, comme l'a rappelé notre collègue Laurence Rossignol. Ce sont bel et bien ces travailleurs du public et du privé qui font tourner le pays et le maintiennent à flot depuis la pandémie. Nous aurions aimé débattre en préambule des facteurs de pénibilité, plutôt que de niveler les droits vers le bas

compter du 1 septembre 2023, les régimes spéciaux de retraites de cinq entités. Cet amendement vise à revenir sur cette suppression. En réalité, les régimes spéciaux concernent non pas l'ensemble des salariés des secteurs concernés, mais uniquement ceux qui ont les conditions de travail les plus pénibles. Ainsi, en 2019, les retraités recevant une pension au titre des régimes spéciaux représentaient environ 6 % de l'ensemble des retraités. Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et d'une supposée universalité est une diversion

qu'elles engendrent, sont particulièrement pénibles. Les régimes spéciaux sont la contrepartie de sujétions particulières. Par ailleurs, les métiers concernés sont essentiels à notre pays de secteurs qui rencontrent des difficultés de recrutement. La mise en cause des régimes spéciaux de retraite renforcera cette carence. Prendre en compte la pénibilité est non pas un privilège, mais une mesure de justice sociale.

sorte, sans aucune négociation, sans aucune compensation et sans aucun accord avec la moindre organisation syndicale. La

beaucoup et il y en a de vrais. Vous avez supprimé l'ISF à un moment où les inégalités de patrimoine augmentaient- rétablissons-le ! Vous avez supprimé la, ce qui fait que le travail est bien plus taxé que le capital- supprimons-la

cette volonté de suppression des régimes spéciaux s'apparente plutôt à une manoeuvre de diversion pour atténuer la seule réalité de cette réforme : le report de l'âge légal, dont tout le monde pâtira incontestablement. Par ailleurs, à l'heure où les secteurs concernés peinent à recruter, la mise en cause de certains régimes spécifiques de retraite est contre-productive.

Fichet, pour présenter l'amendement n° 449. À l'heure où les secteurs concernés sont, pour plusieurs d'entre eux, en manque d'agents et de salariés, la mise en cause des services spéciaux de retraite renforcera cette carence de recrutement.

Selon vous, non seulement il n'est plus possible de prélever le moindre euro supplémentaire sur les grandes entreprises et les grandes fortunes, mais il faudrait même diminuer leur taux de prélèvement.

Pour vous, la vie et le marché se confondent : l'utilité se mesure à la seule valeur commerciale. Avant de vous demander comment améliorer la vie des êtres humains et le sort de la planète qui les nourrit, vous commencez toujours par vous demander à quoi consentiront les puissances de l'argent.

promis, à la Libération, que la retraite serait « non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie ». Vivre décemment jusqu'à son dernier souffle, laisser en paix les corps brisés par l'usure, voilà la grande conquête du XX siècle sur laquelle vous voulez revenir avec cette réforme.

à ses parents dépendants, à ses enfants, à ses petits-enfants, aux vies associative, culturelle, sportive, caritative, démocratique, qui sont essentielles à la vie de notre pays. Voilà ce que vous voulez supprimer !

Certains régimes spéciaux sont des régimes autonomes, qui trouvent leur équilibre dans des niveaux de contribution ou de cotisations délibérément plus élevés que la moyenne.

Mettre fin aux régimes spéciaux, c'est une diversion pour faire oublier la confiscation par le Gouvernement de deux années de retraite à tous les Français. Ne nous laissons pas berner : une vraie mesure de justice sociale et d'équité serait d'appliquer les mesures de prise en compte de la pénibilité à tous les travailleurs et travailleuses qui accomplissent

constat des effets de la pénibilité, un constat du fait que, après des années de dur labeur, les salariés sont « cassés » ? Ceux qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire, ceux qui accompagnent nos aînés, ceux qui construisent nos maisons et nos routes, ceux qui nous transportent midi et soir ne veulent pas que l'on mesure

Jacquin, pour présenter l'amendement n° 808. Cet amendement vise à supprimer l'article 1, car cette réforme des retraites est injuste, injustifiée et inopportune. Elle rencontre l'opposition de la majorité des Françaises et des Français. La suppression des régimes spéciaux ne peut

Ainsi, plutôt que de tout supprimer de manière démagogique, le Gouvernement serait mieux inspiré de retirer sa réforme, de reprendre de véritables négociations avec les partenaires sociaux et d'étudier, profession par profession, l'opportunité de revenir intégralement ou en partie sur certains régimes dits spéciaux. Une bonne réforme des retraites est une réforme qui allie sauvegarde de la répartition et progrès social, pas une réforme qui stigmatise certains et monte les Français les uns contre les autres. Les amendements

Monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'un régime spécial devrait se suffire à lui-même et ne saurait faire appel à personne d'autre que ses clients ou ses agents.

Enfin, les flux futurs de pensions sont déjà intégralement couverts. Alors quoi ? Quelle est la logique de la suppression de ce régime autonome,

je considère que la suppression des régimes spéciaux visés par cet article n'est, sous couvert d'un prétexte d'équité, qu'une diversion pour faire oublier que tout le monde va pâtir du report de l'âge légal de départ à la retraite.

du régime général. Vouloir présenter comme de mauvais élèves des professions qui ont fait, voilà des décennies, le choix de surcotiser constitue une orientation étonnante pour un gouvernement disant défendre le budget de la Nation « à l'euro près Monsieur le ministre, il est temps de comprendre les spécificités de ces professions et d'entendre les difficultés quotidiennes des salariés des industries électriques et gazières, sur lesquels nous devons compter pour rebâtir notre souveraineté énergétique. Il est temps de comprendre les spécificités du régime des salariés de la Banque de France, de celui des clercs de notaire, et de celui des salariés du Cese.

vous avez supprimé les CHSCT et vous voulez déshumaniser encore davantage les entreprises et les métiers ! Il faut supprimer cet article inutile et injuste

permet actuellement. Ces régimes constituent, selon vous, une dépense exagérée qui ne serait plus soutenable par notre système de retraite. En réalité, et vous le savez, les dépenses liées aux régimes spéciaux demeurent contenues en proportion des recettes totales de cotisations sociales.

: conducteurs, agents de station, agents chargés de la maintenance des voies, etc. Non, monsieur le ministre, le départ anticipé de ces personnes n'est ni un privilège hérité de l'ancien monde ni une dépense exagérée, vu la nécessité et la pénibilité et, si les économies engendrées par la suppression de ces régimes sont, pour vous, essentielles, c'est avant tout en raison de leur caractère symbolique d'éradication méthodique des statuts en général

Tout le problème est là : c'est parce que les dégâts du travail n'ont pas été corrigés, parce que l'on a renoncé à améliorer les conditions de travail et parce qu'il n'a même pas été envisagé de prévoir des sources de financement en lien avec la nouvelle donne de la société contemporaine- je pense notamment, comme mes collègues,

prégnants encore que par le passé, les amplitudes horaires et la pénibilité perdurent. Il n'y a donc pas de régime de faveur, il n'y a que la prise en compte de cette dureté, qui abîme. Oui, tous ceux qui font le même travail doivent avoir les mêmes droits et il doit s'agir des meilleurs droits possible, puisque nous sommes pour le progrès social.

pour preuve la sous-déclaration croissante des accidents du travail et des maladies professionnelles. Écoutez, à cet égard, ce que dit la Cour des comptes, qui a récemment signalé la sinistralité hors norme dont souffrent certains secteurs, notamment les métiers du soin et du lien, qui nécessiterait des mesures spécifiques. En réalité, les régimes spéciaux étaient précurseurs d'une juste appréhension du travail et de ses effets sur les travailleurs. Ils ont veillé à maintenir l'équilibre nécessaire entre la vie au travail et la vie en bonne santé L'objectif devrait donc être d'aligner le régime général sur ces régimes, afin de prendre en considération la spécificité des différents métiers, et non l'inverse. J'ajoute qu'il est tout de même extraordinaire de supprimer des acquis sociaux issus, pour bon nombre, d'accords obtenus en 1945, juste après la Libération, au travers d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, sans dialogue, sans négociation avec les partenaires sociaux, sans même l'once d'une compensation ! Vous appelez cela l'équité

pour le Gouvernement, pour vous, monsieur le ministre, de décider de partager largement ces appréciations serait contraire à la séparation des pouvoirs.

En tout cas, nulle générosité, nulle dépense exagérée ici. Vous parlez d'un système qui serait inégalitaire. Oui,

6,4 ans par rapport aux cadres ? Pourquoi n'auraient-ils pas le droit de percevoir, aussi longtemps que les autres catégories professionnelles, leur retraite, celle pour laquelle ils ont cotisé toute leur vie ? Loin de réparer les inégalités au travail, cette Nous devons permettre aux travailleurs de partir à la retraite au moment où leur corps n'est pas usé ; nous le leur devons ! Malheureusement pour eux, votre rhétorique est immuable : vous voulez faire porter aux travailleurs le poids de votre réforme comptable. Ceux qui souffrent déjà aujourd'hui dans leur chair souffriront encore plus demain ; ce sera l'inégalité dans la souffrance. Pour comble, vous simulez une concertation avec les organisations syndicales, sans jamais tenir compte de leurs demandes, de leurs propositions.

« privilégiés »- le mot est lâché -, telle est la vision dogmatique, monsieur le ministre, que votre gouvernement semble avoir des personnes affiliées à un régime spécial de retraite. Je rappelle que les premiers régimes spéciaux ont été mis en place par l'État

Le Gouvernement justifie la suppression des régimes spéciaux par une volonté d'équité, mais il s'agit surtout de diviser les salariés. On le sait bien, depuis Machiavel, diviser pour mieux régner, c'est la solution. En outre, vous faites un choix arbitraire, à la carte, entre les régimes spéciaux qui seront supprimés par cette réforme et ceux qui seront conservés. Alors que plusieurs secteurs concernés pâtissent d'un manque de personnel, la mise en cause des régimes spécifiques de retraite ne fera qu'aggraver leur manque d'attractivité et leur pénurie de personnel. Aussi, plutôt que de défendre un système de retraite adapté à la réalité, notamment à la pénibilité, des métiers, le Gouvernement choisit de détruire ces droits acquis et de niveler ainsi les retraites par le bas. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

ils correspondent à une histoire, mais aussi à un actuel et à un avenir pour beaucoup de salariés. Ce sont des conquêtes sociales qu'il convient de préserver. Nous ne voulons pas nous associer

et des temps de travail, avec une banalisation des emplois précaires, le développement du travail à temps partiel ainsi que la normalisation du travail flexible et irrégulier. À tout cela, il faut ajouter l'insécurité de l'emploi, que de plus en plus de travailleurs perçoivent du fait des multiples restructurations d'entreprises et des licenciements qui vont avec. Depuis plus de vingt ans, la pénibilité déclarée par les salariés est en nette hausse, sur le plan tant physique, avec le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs ou l'exposition à de multiples nuisances, que mental, avec l'exigence d'une vigilance constante, les polyvalences forcées, le raccourcissement des délais ou encore l'exigence d'une réponse immédiate

il convient de s'interroger profondément sur les conditions et l'organisation du travail. Il est grand temps de réduire le temps de travail prescrit et de revenir à la retraite à 60 ans. En effet, si, comme vous, j'accorde une grande importance à l'emploi et au travail, cela ne doit pas se faire au détriment de la santé des travailleurs. Avant de

plus on augmente la part des impôts dans un système par répartition, plus on le remet en cause. C'est pourquoi nous n'avons pas choisi ce dispositif, car nous n'entendons pas remettre en cause le système par répartition.

pionniers furent les premiers à prendre en compte la pénibilité, qu'ils s'appliquent à des métiers en tension, soit du fait d'un manque d'agents, soit pour des raisons d'accidentologie et non de remplacement des agents arrêtés. Vous avez ajouté que ces régimes sont équilibrés, voire excédentaires, et que cette réforme augmenterait les difficultés de recrutement.

Je comprends que les actionnaires de notre pays- mais pas tous -, qui viennent d'encaisser 59,8 milliards d'euros, jugent scandaleux les avantages des chauffeurs de bus de la RATP, dont les conditions de travail sont si favorables que leur employeur ne parvient plus à recruter

(Fonds de réserve des retraites), judicieusement créé par Lionel Jospin pour faire face au papy-boom. Si cela se révélait trop douloureux, de nombreux bénévoles jeunes retraités des Restos du coeur pourraient accueillir ces milliardaires trop taxés mesure permettrait d'économiser deux ans de vie. Enfin, puisqu'il me reste quelques instants, je tiens à dire que je ne comprends pas comment des sénateurs peuvent défendre, au nom de l'équité,

l'idée qu'une entreprise, c'est une communauté humaine dans laquelle les uns et les autres sont solidaires grâce à un statut, des garanties, une protection sociale.

régimes, les travailleurs du régime général étant depuis trop longtemps délaissés au regard de l'évolution des modes de production. Ces régimes spéciaux sont donc des précurseurs en ce qu'ils appréhendent plus justement le travail et ses effets sur les travailleurs.

explication de vote. Je voterai évidemment ces amendements de suppression de l'article 1 pour des raisons de fond,

Pouvez-vous nous expliquer quel sera l'effet direct sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale en 2023, qui sont l'objet même de ce PLFRSS,

conquêtes sociales, cela a déjà été dit, et ont été créés dans le cadre de négociations. Ils sont une juste compensation de conditions de travail difficiles, de perspectives de carrière et d'évolution de salaire parfois plus limitées qu'ailleurs.

On cherche surtout à faire quelques économies de bouts de chandelle sur le dos des travailleurs et à faire diversion pour mieux masquer l'injustice que constitue l'allongement de la durée du travail. Vous cherchez surtout à opposer les Français les uns aux autres pour justifier cette réforme.

au minimum à l'État, voire 50 milliards d'euros si l'on prend en compte certains critères. On voit bien que les économies que l'on cherche à réaliser sur les régimes spéciaux et sur l'ensemble des retraités sont sans commune mesure avec les ressources dont on se prive pour réduire nos déficits.

aggraver ? Nous parlons de plusieurs régimes spéciaux, notamment de celui de la RATP. Quel est l'un des principaux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays ? C'est la crise dans les transports publics, en particulier en Île-de-France.

refusé d'augmenter le versement mobilité des entreprises afin de financer les transports publics en Île-de-France. Elle a par ailleurs refusé d'augmenter, comme elle aurait dû le faire, la participation financière de l'État. Aujourd'hui,

Or, en matière de droit social, la convergence, toute l'histoire du droit social le montre, c'est la généralisation progressive des dispositions les plus protectrices. Cela n'a jamais été le contraire ! Vous voulez la retraite

J'ai écouté avec attention la rapporteure générale et le rapporteur Savary, puis j'ai lu l'amendement n° 2057 de M. Retailleau et d'un certain nombre de ses collègues. Depuis, je ne m'y retrouve plus

qui prétendent ici, aujourd'hui, agir au nom de l'égalité. Cela nous a été dit. La suppression proposée vise en réalité un alignement vers le bas et, finalement, la destruction de ce qui peut être qualifié de droit visant à une plus grande justice sociale. Il faut plutôt voir ces régimes spéciaux comme des modèles. Ils ont servi de point d'appui à la mise en place d'une couverture vieillesse généralisée. pouvons encore nous en inspirer pour continuer à améliorer le régime général d'assurance vieillesse, notamment par la prise en compte des spécificités des différents métiers, dont la nature évolue, tout comme la pénibilité qui les caractérise. Je voterai donc l'amendement visant à maintenir

pas des privilèges : ils représentent l'héritage de régimes fonctionnant sur la base d'une solidarité interprofessionnelle ou propre à une entreprise. Ils prévoient des règles de départ à la retraite spécifiques, car ils prennent en compte une pénibilité spécifique à laquelle les travailleurs qui cotisent

vos interventions et de connaître votre point de vue sur ces amendements de suppression et sur la remise en question des régimes spéciaux. Là encore, je considère que le débat est tronqué, puisque nous ne connaissons pas votre point de vue sur ces amendements.

assemblée ? Je comprends pourquoi vous vous entêtez à garder confidentielle la note du Conseil d'État : cela tient certainement à la fragilité de la place de cet article dans le texte ... J'ai parlé tout à l'heure de la paresse, voire de la torpeur qui avait gagné les rangs de la majorité sénatoriale.

Et vous leur envoyez le message que la pénibilité n'existe pas ! Ceux qui bénéficiaient d'une prise en compte de celle-ci au travers de leur régime de retraite vont perdre ce qui n'était pas un avantage, mais une juste prise en compte de leur engagement professionnel. Si nous voulons réhabiliter le travail et réduire les tensions dans un certain nombre de secteurs, ce n'est pas en alignant par le bas les acquis sociaux que l'on y arrivera. C'est la raison pour laquelle il faut maintenir ces cinq régimes dits spéciaux et surtout engager des négociations avec les partenaires sociaux sur la pénibilité. Mais ce mot a été rayé du projet de loi et ne fait l'objet d'aucun article

aux risques au fil de la carrière. Selon la pénibilité, on peut bénéficier d'une majoration de la durée de service, qui se traduit par une anticipation de l'âge du départ à la retraite.

comme à la RATP, mais aussi réduire la semaine de travail. Non, monsieur le rapporteur Savary, il ne suffit pas de faire silence sur la dureté de ces métiers pour améliorer leur attractivité. Déjà, il n'y a plus d'aides-soignants et d'aides à domicile pour entrer dans nos services. La solution, ce n'est pas les exosquelettes, mais la réduction du temps de travail.

négligez les salariés concernés par ces régimes spéciaux alors que les cabinets de conseil s'engraissent régulièrement sur les carences, les défaillances et les incohérences de votre gouvernement.

Il faut également, pour le développement économique et social, que cet article, injustifié, soit supprimé.

non seulement pour défendre les régimes spéciaux, mais parce que je pense qu'autre chose se joue dans cette affaire. Voilà plusieurs années que j'observe les libéraux faire des

Plus notre pays est fragmenté, plus vous incitez nos concitoyens à chercher les responsables de leurs souffrances à côté d'eux, au plus proche d'eux. En fait, c'est une méthode assez facile, qui consiste à faire croire au salarié que, s'il n'est pas assez payé, c'est à cause du chômeur ; au chômeur que, s'il n'est pas assez indemnisé, c'est à cause de celui qui est au RSA ; et à ce dernier que,

parce que les gens perdent en identité nationale, mais parce que le progrès social et le progrès républicain, qui faisaient le ciment du sentiment national et de la cohésion des citoyens dans la République, ne sont plus au rendez-vous. Avec

Depuis le début de ce débat, on nous explique que cette réforme répond à des exigences de nature budgétaire et comptable pour rééquilibrer un système de retraite par répartition supposément déficitaire. Pourtant, il apparaît qu'en supprimant le régime spécial de la RATP, vous allez créer un déficit supplémentaire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Christophe Rolin, le directeur de la caisse de retraite de la RATP,

Le contribuable, lui, sera contraint de compenser l'aggravation du déficit : celui-ci s'élève à 780 millions d'euros par an aujourd'hui, avec votre réforme, la note passera à 1,2 milliard d'euros par an d'ici quatre ans. Chez les électriciens et gaziers,

et le taux de service est de 100 % : il faut donc savoir raison garder. Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et d'une prétendue universalité est une diversion, pour faire oublier que tout le monde va pâtir du report de l'âge légal. La justice sociale et l'équité consisteraient justement à appliquer des mesures sérieuses de prise en compte de la pénibilité à l'ensemble des travailleurs qui accomplissent des travaux pénibles, plutôt que de niveler par le bas. Voilà pourquoi il faut absolument supprimer cet article.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.